notre séance se déroule dans les conditions de respect des règles sanitaires mises en place depuis le mois de mars. L'hémicycle fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection avant et après chaque séance, et les micros seront désinfectés après chaque intervention. J'invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité. Les sorties de la salle des séances devront exclusivement s'effectuer par les portes situées au pourtour de l'hémicycle. Je rappelle également que les orateurs s'exprimeront depuis leur place, sans monter à la tribune. Notre séance s'organisera en trois temps : après la déclaration du Gouvernement, la parole sera donnée à un orateur de chaque groupe

la crise sanitaire que nous vivons et qui frappe le monde entier a une dimension inédite. Cette situation, qui est exceptionnelle par sa gravité, par les deuils et les sacrifices qu'elle a imposés à beaucoup de nos concitoyens, nous oblige à apporter des réponses adaptées. Nous avons le devoir d'envisager toutes les solutions possibles et de mobiliser toutes les ressources pour mettre un terme à cette situation. La volonté- et l'obligation -du Gouvernement est que son action s'inscrive dans ce domaine, sans exception possible, dans le cadre des valeurs de notre démocratie, c'est-à-dire le respect de l'État de droit et des libertés individuelles. C'est en nous conformant à cette exigence que nous pourrons conserver la confiance de nos concitoyens. Les services numériques offrent évidemment d'immenses opportunités, vous le savez. Durant la crise, ils ont démontré leur intérêt et leur potentiel dans le domaine des consultations en télémédecine, qu'il s'agisse également du télétravail ou bien de l'école à distance. Encore faut-il que ces outils numériques soient utilisés dans un cadre protecteur et respectueux des droits de chacun. Cet encadrement a été bâti, adapté et perfectionné progressivement, afin de garantir à chaque personne la protection de ses droits fondamentaux, ainsi que le respect de sa vie privée et de ses données à caractère personnel. La France, vous le savez puisque vous avez été des acteurs dans ce domaine, a toujours été à l'avant-garde de la protection des données et de la garantie des libertés individuelles dans ce domaine. La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 nous a permis d'être le premier pays en Europe à se doter d'un texte général, fondateur, protégeant les données à caractère personnel. Et c'est cette loi qui a créé la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), dont nous savons aujourd'hui encore combien elle est indispensable. L'Union européenne, pour sa part, a élaboré, d'ailleurs sous l'impulsion de la France, entre autres, un cadre juridique harmonisé et protecteur pour les citoyens européens, pour l'utilisation de leurs données à caractère personnel. Ainsi, la directive Vie privée et communications électroniques du 12 juillet 2002 permet de garantir la protection de la vie privée lorsque des correspondances empruntent des moyens de communication électroniques.

Ces textes nationaux et européens n'interdisent d'aucune manière l'utilisation des données personnelles dans le cadre d'une stratégie sanitaire, mais ils ont posé de grands principes auxquels doit se conformer tout traitement de données à caractère personnel. Ces grands principes constituent des garanties pour le respect de notre vie privée et de nos libertés individuelles. Trois d'entre eux, définis à l'article 5 du RGPD, constituent une base, un socle essentiel qui doit être ici mentionné. Le premier principe, c'est celui dit « de la limitation des finalités ». Principe cardinal de la protection des données à caractère personnel, il établit que ces dernières ne doivent être utilisées que pour pour un objectif précis et déterminé à l'avance. Selon les termes mêmes du RGPD, le traitement doit répondre à une finalité déterminée, explicite et légitime. Déterminée, parce qu'il n'est pas possible de collecter des données sans but ou à des fins préventives ; explicite, parce que les personnes concernées doivent savoir pourquoi et comment leurs données sont traitées ; légitime, parce que le traitement doit être en rapport avec l'activité de celui qui en

l'exécution d'un contrat ou l'exécution d'une mission d'intérêt public- et ce sera le cas ici. Enfin, le troisième principe est celui dit « de minimisation des données » ou « principe de proportionnalité Cela signifie que l'on ne peut traiter que les données pertinentes et strictement nécessaires au regard de la finalité du traitement. Ces principes ont été respectés pour chacun des outils numériques mis en place par le Gouvernement pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19, qu'il s'agisse de Contact Covid ou du système d'information national de dépistage, le Sidep, deux traitements autorisés par le décret du 12 mai dernier. Ils permettent d'identifier les personnes infectées, les personnes qu'elles sont susceptibles d'avoir contaminées les chaînes de contamination. Ces traitements visent également à assurer la prise en charge sanitaire et l'accompagnement des personnes atteintes du virus ou susceptibles de l'être, ainsi que la surveillance épidémiologique du virus. L'application StopCovid a respecté les mêmes principes posés par le RGPD. Elle complète les outils développés dans le cadre de la stratégie de déconfinement progressif que le Gouvernement a souhaité mettre en place. Ces trois dispositifs, qui utilisent des données à caractère personnel et qui s'inscrivent donc dans une politique sanitaire globale, ont été soumis à l'avis de la CNIL, qui a donné un avis favorable. Cette application a d'ailleurs fait l'objet de deux avis de la CNIL : l'un du 24 avril et l'autre du 25 mai. La CNIL s'est félicitée dans son dernier avis que ses premières recommandations aient été suivies par le Gouvernement.

StopCovid répond aux exigences posées par notre droit et, me semble-t-il, apporte les garanties nécessaires au respect de la vie privée et des libertés individuelles. Cela résulte à la fois de ce qu'est l'application StopCovid et de ce qu'elle n'est pas.

d'emblée primordial de préciser qu'il ne s'agit en aucun cas de procéder à la géolocalisation des personnes ou à un suivi intrusif de leurs déplacements.

Nul ne sait où la personne est allée ni où elle a rencontré d'autres personnes susceptibles d'avoir été infectées ; on sait seulement que des personnes ont croisé l'utilisateur de l'application. StopCovid n'a d'ailleurs pas non plus vocation à permettre un quelconque fichage des Français ou à contrôler leur respect des mesures sanitaires. Le décret créant cette application sera très clair, en précisant expressément ce à quoi elle peut servir. J'ai dit ce que n'était pas StopCovid ; j'ajouterai quelques mots maintenant sur ce qu'est cette application. Il apparaît nécessaire, dans le cadre de la stratégie globale de déconfinement du Gouvernement, non seulement d'être capable d'identifier ceux que l'on appelle les « cas contacts », qui sont les proches des personnes infectées, connus de ces dernières, mais aussi d'être en mesure d'alerter tous les autres, ces inconnus croisés dans les transports ou dans les magasins et qui ont pu être contaminés sans le savoir. Il s'agit ainsi de juguler aussi rapidement que possible et aussi efficacement que possible les chaînes de contamination. C'est là l'objectif de cette application. Et c'est donc bien sur le fondement de l'exécution d'une mission d'intérêt public d'une mission d'intérêt public que ce traitement sera mis en oeuvre, sous la responsabilité du ministère des solidarités et de la santé. De nombreuses autres garanties entourent ce traitement, conformément aux préconisations de la CNIL. J'en citerai quatre. l'utilisation volontaire de cette application. À chaque étape, le consentement des personnes est requis et leur choix est garanti. Le téléchargement de l'application résulte d'une démarche volontaire de l'utilisateur ; son installation est est libre et gratuite ; les fonctionnalités ne pourront être activées que si l'utilisateur le souhaite ; la désinstallation sera possible à tout moment. Si un test nasopharyngé permet à l'utilisateur de savoir qu'il est potentiellement contaminant, il ne le notifiera dans l'application que s'il le souhaite. Recourir ou non à l'application est donc un choix que chacun d'entre nous pourra faire. Notre liberté est ainsi préservée et garantie. Précision capitale pour que cette liberté soit garantie : aucune conséquence négative n'est attachée au choix de ne pas recourir à cette application. L'accès aux tests et aux soins, la liberté d'aller et de venir, l'accès aux transports en commun ne sont pas conditionnés à l'installation et à l'utilisation de l'application. Il ne saurait non plus y avoir de conséquences sur la vie professionnelle. De même, ni son installation ni son utilisation ne donnent droit à aucun droit ou avantage spécifique. Le consentement est donc libre, conformément à notre droit national et à la réglementation européenne que j'ai citée tout à l'heure. que j'ai citée tout à l'heure. La deuxième garantie, c'est la pseudonymisation. L'installation de l'application ne requerra pas la fourniture de données directement identifiantes comme le nom ou l'adresse. Seuls des pseudonymes éphémères seront utilisés, ni l'État ni personne d'autre n'aura accès à une liste de personnes diagnostiquées positives ou à une liste des interactions sociales entre les utilisateurs. La troisième garantie est la conservation des données pour une durée extrêmement limitée. Les données ne pourront être gardées que pendant la durée de fonctionnement de l'application.

insiste. Sa mise en oeuvre est fixée à six mois, une durée qui correspond à celle qui est prévue pour les traitements Contact Covid et Sidep, l'application n'ayant en réalité d'utilité qu'en lien avec le cadre plus général de conduite des états sanitaires. Plus encore, les historiques de proximité ne pourront être conservés que quinze jours, durée strictement nécessaire au regard de la durée d'incubation du virus. Plus important encore, l'utilisateur pourra à tout moment demander la suppression de ces données tant de son ordiphone que du serveur central. Enfin, la dernière garantie est la transparence. L'application StopCovid s'inscrit dans une démarche de transparence. Les utilisateurs seront informés des principales caractéristiques du traitement et de leurs droits au moment de l'installation de l'application. StopCovid respecte donc strictement la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi que les préconisations de la Commission européenne, du Comité européen de la protection des données et de la CNIL,

non identifiante et transparente. Toutes les garanties me semblent donc prises pour que la vie privée des Français soit respectée.

d'ériger un État policier, contrôlant les faits et gestes de nos concitoyens. À juste titre, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) souligne qu'« il s'agit de sujets de préoccupation majeurs dans une société démocratique, nécessitant une transparence accrue et des garanties suffisantes pour pallier les risques d'atteinte transversale aux droits et libertés fondamentaux

le combat n'est pas terminé, et nous devons étudier tous les outils permettant de vaincre le virus. Le débat qui nous réunit ce soir est celui de la pertinence et de la juste mesure. la première question est la suivante : l'application StopCovid est-elle efficace ? De nombreuses études épidémiologiques montrent l'intérêt que présentent, pour les autorités sanitaires, les applications

vote que vous avez émis il y a quelques semaines, le suivi des contacts est réalisé manuellement, au moyen d'une enquête auprès de la personne malade, qui transmet la liste des personnes avec qui elle aurait été en contact et celle des lieux publics qu'elle a visités durant sa période de contagiosité. L'action de traçage n'est pas nouvelle : cette méthodologie est largement utilisée en veille sanitaire, pour bon nombre de pathologies infectieuses à transmission interhumaine.

Ces équipes d'anges gardiens sont indispensables pour intervenir rapidement et casser les chaînes de contamination. Les dernières données le prouvent : près de 45 % des transmissions du virus se font à partir de personnes asymptomatiques.

L'Académie de médecine a émis un avis favorable à l'utilisation d'une application de type StopCovid, dans le cadre du déconfinement. Ce dispositif permet une participation active de la population à la lutte contre la pandémie,

vie privée. Pour concilier ces deux protections, il faut assumer la transparence. Vous le savez, StopCovid a été développé sous la supervision du ministère des solidarités et de la santé et du secrétariat d'État chargé du numérique. Dans un avis datant d'avril dernier, le Conseil national de l'ordre des médecins a précisé ses recommandations en matière d'utilisation du numérique dans la période d'épidémie. Ces préconisations ont été suivies. L'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) a été chargé de développer un prototype d'application et d'instruire les différentes questions techniques. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a quant à elle été sollicitée pour garantir la résilience et la sécurité des solutions étudiées.

La transparence est une clé essentielle de StopCovid. La protection de la vie privée est un principe avec lequel nous ne transigerons pas. L'application StopCovid ne doit pas passer pour autre chose que ce qu'elle est fondamentalement : un simple outil de lutte contre une épidémie redoutable ; un outil efficace et- j'en suis profondément convaincue -un outil légitime.

: le site « mesconseilscovid.sante.gouv.fr », qui permet à chacun de nos concitoyens de bénéficier d'informations utiles pour se protéger et pour protéger les autres. Cet outil intervient en amont de l'entrée dans le parcours de soins. dispense sont personnalisés selon la situation médicale, familiale, professionnelle et géographique de l'utilisateur, sans stockage de données sur un serveur central.

Afin de soutenir ce formidable élan et d'accompagner à la fois les citoyens, les professionnels et les établissements de santé dans leurs choix d'outils numériques, le Gouvernement a lancé une plateforme de référencement, véritable guichet de l'innovation numérique dédié

Il s'agit donc d'une première, mais probablement pas d'une dernière. Ce que nous savions, et que le confinement a confirmé de manière paroxystique, c'est que le numérique est devenu la colonne vertébrale de notre économie, de notre société et même de nos institutions. cette dorsale a ses propres déterminants et ses propres règles, que le champ législatif et l'action politique méconnaissent trop souvent. Les langages du droit et de la loi ont, à nos yeux, une noblesse que le code informatique n'a pas encore, même s'il tend souvent à les supplanter.

Le résultat d'une notification positive est d'ailleurs en ligne avec la doctrine relative aux cas contacts : une fois notifié, vous devrez vous isoler, prendre contact avec un médecin et, le cas échéant, être testé.

comme le prouvent de nombreux travaux scientifiques, ces heures et ces jours sont décisifs : plus de la moitié des contaminations sont le fait de personnes en période d'incubation ou asymptomatiques. Elles contaminent leurs proches et d'autres individus sans le savoir. Dans ce contexte, StopCovid n'est en aucun cas la solution magique. Mais l'application apporte une réponse à ces difficultés. Elle offre un complément utile et nécessaire au travail, central, des équipes d'enquête sanitaire.

Si nous voulons éviter une seconde crise sanitaire, nous devons nous en donner les moyens. D'un point de vue sanitaire, l'application StopCovid, dûment encadrée, doit faire partie d'une stratégie nationale de contrôle de l'épidémie. »

Certains redoutent une société de la surveillance, dénoncent le et la géolocalisation, demandent à ceux de leurs proches qui téléchargeraient l'application de les supprimer de la liste de leurs contacts. Je veux les rassurer : de tout cela, il n'est en La seule technologie utilisée est le Bluetooth. La seule information disponible est la notification anonyme reçue, et reçue par vous seul, lorsque vous avez été en contact prolongé avec une personne testée positive

convaincu : les nouvelles technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises par essence. Il nous revient de bâtir les contre-pouvoirs et les institutions qui nous protègent des tentations et des dérives que peuvent

de spécialistes de la santé, des questions d'éthique et du numérique, mais aussi de parlementaires. Ce comité pourra diligenter tous les audits nécessaires sur le serveur central, afin de vérifier que celui-ci fait bien ce que le Gouvernement dit qu'il fait,

à évaluer, auditer et surveiller l'ensemble des outils numériques de traçage mis en place par le Gouvernement, dont StopCovid. C'est bien simple : l'intérêt du Gouvernement et des autorités sanitaires, c'est de faire la transparence totale sur le fonctionnement de cette application,

La politique, le droit, la vie, tout est affaire de proportions. Ce qui compte, c'est l'équilibre. Telle est la question en balance : y a-t-il un plus grand risque sanitaire, social, économique, voire démocratique que la perspective du reconfinement ? C'est cette proportionnalité qui a conduit le Comité national pilote d'éthique du numérique, au sein du Comité national consultatif d'éthique, à insister sans délai sur l'importance d'une telle application de suivi numérique de contacts, dont le contrôle souverain doit être garanti aux citoyens français, voire européens, dès lors que l'on aura statué sur ses qualités éthiques.

sûr, il a des échos et des ramifications européennes, mais ne nous y trompons pas : ce qui tiendra, demain, derrière une petite icône sur chaque téléphone est le fruit de milliers d'heures de travail et de nuits courtes, en faveur d'un projet emblématique du savoir-faire des chercheurs, des industriels et des entrepreneurs français.

Ce refus n'a rien de dogmatique. Il n'est pas opposé, en soi, parce qu'il s'agit d'Apple et de Google ; mais parce qu'une grande entreprise, si performante et innovante soit-elle, n'a pas à contraindre les choix de politique sanitaire d'une nation souveraine ; parce que, pour garantir la sécurité des données des Français et l'efficacité sanitaire du dispositif, la France a fait le choix de l'indépendance. Nous ne sommes pas au bout du chemin, loin de là ; vous pourriez du reste décider que la route s'arrête là.

À l'heure où le monde du numérique et, parfois, le monde tout court, tend à être dominé par une poignée d'entreprises quasi oligopolistiques, c'est cette même alliance de la recherche, des grandes entreprises, des start-up et des institutions qui doit permettre à la France de tirer son épingle du jeu et de conserver son indépendance sanitaire et technologique.

cette histoire. Le progrès, aujourd'hui, n'a plus si bonne presse. Des OGM à la 5G, de l'intelligence artificielle aux cellules CAR-T, une partie de la France n'ose plus regarder l'innovation en face. Sondage après sondage, le pessimisme semble gagner du terrain. La science recule au rythme où progressent les fausses informations et les prophètes autoproclamés. Maintenant, c'est de la lévitation ... Bien sûr, le réchauffement climatique est là pour nous rappeler chaque jour que le progrès n'est pas bon en soi, qu'il doit être maîtrisé et piloté. un pays qui a peur d'innover, qui se défie de ceux qui prennent ce risque, qui fait du principe de précaution l'alpha et l'oméga de tous ses débats, est un pays qui se contente

Mais l'espoir n'a jamais fait une stratégie. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que tous les outils soient déployés, dès lors qu'ils respectent nos valeurs, pour mieux combattre l'épidémie.

Pour autant, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les développements du projet d'application StopCovid. En effet, j'en suis également convaincu : on ne peut pas nier la nécessité de sortir au plus vite, et dans les meilleures conditions, de cette pandémie qui a déjà fait beaucoup de dégâts. Je regrette profondément que le projet qui regroupait 135 chercheurs issus de 8 pays européens ait achoppé sur l'opposition entre centralisation et décentralisation invoquée par nos amis suisses. l'irruption des sociétés Apple et Google, qui se sont alliées sur ce sujet d'une manière un peu improbable, mais sûrement pas innocente, ... Et surtout opportuniste ! ... a contribué à faire voler en éclats le consensus européen. J'approuve donc la volonté du Gouvernement de faire en sorte que ces sociétés ne puissent pas s'approprier encore un peu plus nos données. J'espère que les talents que vous avez réunis autour de l'Inria dans le cadre d'un partenariat public-privé public-privé ont élaboré une application dans laquelle nous pourrons avoir confiance, mais qui permettra aussi l'interopérabilité avec les pays européens. Dans la mesure où vous serez en capacité de nous garantir la limitation dans le temps de l'usage de dans la mesure où vous pouvez nous garantir que cette technologie reposera sur le volontariat et l'anonymat des personnes, dans la mesure où cette pratique sera assortie d'une politique de tests massive indispensable, politique qui n'a pas encore été pratiquée jusqu'à présent, je voterai en faveur de la mise en oeuvre de cette technologie, car l'essentiel est que nous puissions sortir rapidement de cette pandémie dont nous n'avons pas fini de payer les dégâts humains, sociaux et économiques. Soyez toutefois certain

du Parlement, mais soyons francs : quelle valeur accordez-vous au vote du Sénat ? N'est-il pas symbolique ? Restera-t-il, comme le vote sur le plan de déconfinement, lettre morte ? ? La réalité est que nous n'avons pas notre mot à dire, puisque la validation, déjà acquise par la majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale, vous suffit pour clore le parcours semé d'embûches de cette application. Un renoncement à sa mise en oeuvre aurait été préférable, d'autant que, même si vous vous montrez catégorique quant aux précautions prises en matière de respect des libertés publiques, de nombreuses questions d'ordre éthique, politique,

Pour ce qui est des difficultés techniques, on peut s'interroger sur la technologie Bluetooth choisie, qui, bien qu'elle permette d'éviter la géolocalisation, pose tout de même de nombreux problèmes de sécurité. Selon les spécialistes, cette technologie est une véritable passoire, maillon faible des smartphones par lequel les pirates peuvent pénétrer dans nos mobiles. Par ailleurs, alors que vous estimez avoir eu l'assentiment de la CNIL, qui pour sa part a effectivement noté le respect des principes fondamentaux, vous omettez de relever une des failles soulevées dans son avis rendu public cette semaine en l'état du projet de décret- car nous n'avons pas à cette heure la totalité du dossier-, la commission estime que les droits d'accès, d'effacement ou d'opposition ne s'appliquent pas. Or ils le devraient, dès lors que le traitement est basé sur le volontariat.

rappelle sur leur site relatif au traçage numérique un principe essentiel en sécurité informatique : l'innocuité d'un système ne doit en aucun cas être présumée en comptant sur l'honnêteté de certains de ses acteurs. Ils alertent sur le fait que, outre les pouvoirs publics, d'autres acteurs collectifs ou individuels sauront tirer profit des propriétés de ces systèmes, comme autant de failles mettant à mal les libertés individuelles. En outre, parmi les craintes de glissement subsiste l'idée paradoxale que l'usage d'une application pourrait être volontaire, mais que son non-usage pourrait toutefois vous être reproché. Dites-moi quel usage en fera par exemple tel ou tel employeur ou organisme privé, et alors du consentement de celles et ceux qui se verraient fortement incités à l'installer ? J'en viens donc aux questions éthiques. L'implication de grands groupes privés dans la mise en oeuvre de l'application et, demain, dans son développement, n'est pas pour nous rassurer, sans parler des bénéfices que cela générera par voie publicitaire pour les Gafa, qui sont incontournables sur le marché. Ainsi, dans une tribune du du 25 avril, trois spécialistes du numérique alertaient sur l'ombre d'intérêts privés et politiques qui pèseraient sur le projet StopCovid : « Le Le modèle de gouvernance qui accompagnera StopCovid sera manifestement concentré dans les mains d'une poignée d'acteurs étatiques et marchands. Une telle verticalité n'offre aucune garantie contre l'évolution rapide de l'application en un outil coercitif, imposé à tout le monde. » » Vous vous appuyez aujourd'hui sur les demandes des médecins et des épidémiologistes, qui seraient tous favorables au développement de cette application. Je pourrais en citer qui y sont opposés, mais le Parlement est seul juge

concernant les moyens des hôpitaux. Cette application n'assure pas l'équilibre entre liberté individuelle et efficacité sanitaire. Elle ouvre la voie à des usages futurs et à l'adoption de dispositifs très intrusifs. Nous sommes face au risque de créer un précédent. Ce qui paraît acceptable pour StopCovid le sera demain dans d'autres domaines et pour d'autres finalités. Lesquelles

traçage, pistage, suivi des contacts, historique des rencontres, signalement des contaminations : à ces mots, certains ont pu se demander si Big Brother n'était pas en train de faire son entrée dans le domaine de la santé, ... C'est Si l'intitulé de notre débat vise les innovations numériques dans la lutte contre l'épidémie, il n'aura échappé à personne que la star en la matière est bien l'application StopCovid. sa pertinence, aux risques qu'elle emporte et à son fonctionnement on fait couler beaucoup d'encre. Deux points principaux cristallisent les débats : l'atteinte possible aux libertés individuelles, et l'efficacité sanitaire d'une telle application. À l'ère du traçage numérique, il est parfaitement compréhensible, et peut-être même sain, qu'une application visant à retracer les rencontres entre les individus suscite des interrogations. Plusieurs pays plus ou moins démocratiques travaillent à des dispositifs plus ou moins liberticides. Certains d'entre eux s'appuient sur la géolocalisation des individus, d'autres imposent l'installation de l'application, d'autres encore s'en remettent à Google et à Apple. Le Gouvernement a fait l'effort, malgré les pressions, de développer une solution française en refusant d'accroître la dépendance de la France à l'égard des Gafam. Nous espérons qu'il s'agit des premiers pas vers une souveraineté numérique, si essentielle à nos yeux. L'approche en code source ouvert nous semble également une bonne idée. Elle permettra, d'une part, de vérifier que l'application est conforme aux annonces, et, d'autre part, d'augmenter le niveau de sécurité de l'application. Il faudra veiller en particulier à ce que personne n'ait accès aux identifiants des malades ou à des cas contacts, et à ce que personne ne soit contraint d'installer l'application. Nous nous réjouissons que le Gouvernement soit parvenu à proposer, en un temps très court, une solution qui est probablement la plus respectueuse possible des libertés. La CNIL a rendu hier un nouvel avis sur la question, dans lequel elle indique que ses recommandations ont été entendues. Elle a précisé à cette occasion que la création de StopCovid avait respecté le concept dit « de protection des données dès la conception Certains ont déploré cette approche libérale, en faisant rimer autorité avec efficacité. Mais nous ne devons pas sacrifier les principes qui sont les nôtres : les libertés individuelles sont essentielles à notre démocratie ; elles ne sont pas une option. Si des restrictions apparaissent nécessaires, nous devons veiller à ce qu'elles soient les plus limitées possible. La responsabilité des individus, à laquelle notre groupe croit beaucoup, implique d'ailleurs que ces derniers disposent de leur liberté de choix. Aussi, si elle n'est pas obligatoire, StopCovid est-elle encore utile ? Études à l'appui, nous avons entendu des voix s'élever pour affirmer qu'elle serait en fait dépourvue d'effets. Nous n'avons pas de telles certitudes. Vous avez, madame la garde des sceaux, madame, monsieur les secrétaires d'État, rappelé les situations dans lesquelles les enquêteurs sanitaires sont démunis. C'est notamment le cas dans les zones urbaines denses, mais aussi dans les transports en commun. Nous ne connaissons pas l'identité des personnes que nous croisons dans la rue, et c'est heureux. Nous ne savons pas avec qui nous voyageons dans les trains et les métros. Il est donc impossible de prévenir ces personnes si nous tombons malades. Les enquêteurs sanitaires ne le pourront pas non plus. À ce jour, seule une application permet de remédier à ces cas de figure. Les garanties apportées par le Gouvernement nous semblent suffisamment solides. Nous serons cependant très attentifs à l'utilisation de StopCovid. La technologie n'est pas une panacée : elle est utile dans la lutte contre l'épidémie, mais elle ne nous dispensera jamais de l'humain. Nous sommes ainsi particulièrement vigilants quant aux moyens dont disposent les enquêteurs sanitaires. Il est indispensable qu'ils soient suffisamment nombreux pour retrouver et accompagner l'ensemble des personnes susceptibles d'avoir été infectées. La France continue de vivre avec le risque de Covid-19. Dès lors qu'ils ne contreviennent pas à nos principes, tous les outils qui contribueront à faire reculer le virus bénéficieront du soutien du groupe Les Indépendants. Mes chers collègues, la pire des privations de liberté que nous ayons connue, c'est le confinement. Les outils qui, dans le respect de nos principes démocratiques, pourront éviter un nouveau confinement bénéficieront donc du soutien du groupe Les Indépendants.

le débat et le vote de ce soir n'ont d'existence que par la volonté de l'exécutif de consulter le Parlement sur la mise en place d'une application numérique de traçage social appelée « StopCovid Ce débat et ce vote revêtent à mes yeux un caractère beaucoup plus politique et philosophique que technique et juridique. Si l'on ne peut négliger le contexte dans lequel nous débattons, alors qu'un virus a tué 30 000 de nos compatriotes et mis notre économie à genoux,

conforme au droit national et communautaire en tenant compte des deux avis de la Commission nationale informatique et libertés. Je sais aussi que vous vous employez à rassurer ceux qui, comme moi, ont de fortes réserves sur ce dispositif. au sein du Parlement de notre République, où s'exprime la volonté populaire, je dois vous dire que lorsque je fais rationnellement le calcul des coûts et des avantages de cette application, je lui trouve tellement de défauts et si peu de mérites qu'il m'est impossible, comme à un certain nombre de membres de mon groupe, de vous donner mon accord. Tout d'abord, sur le plan des principes, je combats fermement cette idée du « solutionnisme » technologique à tous crins, qui peut voir les principes de protection de la vie privée comme des freins au progrès,

n'a pas déjà entendu dire que la loi de 1978, la CNIL ou le RGPD étaient des contraintes trop lourdes, qui empêchent la croissance de la nouvelle économie ? Qui n'a jamais entendu dire que notre cadre législatif français et européen nous privait de toute perspective de victoire dans la compétition internationale Monsieur le secrétaire d'État, vous nous demandiez ce matin en commission des lois quel pourrait être le gain politique recherché par la mise en oeuvre de cette application. À la lumière de ce que je viens de vous dire, je me pose également la question, mais je suis sûr que je n'y apporterais pas les mêmes réponses que vous. vous. En termes de temporalité, ensuite, si cette application avait dû être mise en oeuvre, en toute logique, elle aurait dû l'être comme un outil de confinement, au moment même où nombre de nos libertés étaient si lourdement atteintes liberté d'aller et de venir, la liberté du commerce et de l'industrie, le droit de vote. Ce qui aurait pu être une application de confinement est mis en oeuvre environ un mois après le début du déconfinement, ce qui lui donne beaucoup moins d'efficience, alors que l'on sait que l'acceptabilité sociale risque d'en être trop faible. de relayer ici l'inquiétude de certains maires et présidents de collectivités locales, qui s'étonnent que l'on évoque un consensus de leurs associations à ce stade du débat. Enfin, je ne puis passer sous silence la question de la souveraineté numérique. Monsieur le secrétaire d'État, vous nous avez annoncé il y a quelques semaines une application souveraine et européenne. On nous a vanté le travail collaboratif entre l'Inria, la Fraunhofer Gesellschaft en Allemagne et l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. L'argument était particulièrement vendeur et convaincant. Je me suis même demandé comment je pourrais ne pas soutenir une telle initiative, qui unissait les instituts de recherche publics européens

cette application nous fait à mes yeux franchir deux lignes rouges. La première est l'expérimentation massive d'une application de traçage social avec la construction d'une architecture numérique centralisée.

Nous ne sommes qu'au début d'un basculement. Des digues auront rompu, car les nouvelles fonctionnalités offertes ouvriront naturellement le champ à d'autres finalités.

de La Boétie : « Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir : il sert si bien, et si volontiers, qu'on dirait

la lutte contre le virus devra concentrer ses efforts et ses moyens sur la façon dont nous pouvons casser les reins de cette épidémie.

de lutter contre une épidémie et de sauver des vies, mais pas au prix du reniement de ce que nous sommes et de nos propres valeurs démocratiques et républicaines. Il y a deux mois- le 8 avril, ce n'était pas hier -j'ai écrit au Président de la République pour lui demander deux types de garanties. La réponse m'est parvenue seulement ces dernières heures, mais je sais qu'il y a loin de l'Olympe à la terre.

Mais ce serait surtout abdiquer notre statut de citoyens pour un statut médiocre de consommateurs dociles, ma chère Catherine Morin-Desailly, au sein d'une colonie numérique américaine.

Nous vous en remercions et nous pouvons d'ores et déjà noter que le débat sur cette question sensible se déroule, du moins dans cette assemblée, dans un climat plutôt apaisé. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, nous avons eu de nombreux débats moins sereins.

La solution que vous nous proposez poursuit des objectifs utiles, et il faudrait être de mauvaise foi pour affirmer que rien n'est fait pour résoudre les différentes problématiques auxquelles elle est confrontée. J'aborderai toutefois plusieurs des dilemmes qui se sont présentés à vous, vous avez fait des choix techniques discutables qui ne peuvent pas tous être balayés d'un revers de la main. Fallait-il, par exemple, opter pour une architecture centralisée ou pour des données décentralisées sur les téléphones des utilisateurs ? Je ne suis pas spécialiste de sécurité informatique, mais on peut comprendre que ces deux solutions ont des arguments en leur faveur. Vous avez retenu une ossature centralisée, suffisamment sécurisée d'après vous. Nous pouvons l'entendre, même s'il subsiste des doutes sérieux sur l'inviolabilité du fichier centralisé. Par ailleurs, la solution décentralisée permet souvent de créer plus de confiance chez les utilisateurs. Le choix de cette solution vous a fait perdre la participation- loin d'être anecdotique -, de nos voisins allemands- ce n'est pas à vous que j'apprendrai leur exigence en matière de protection des données. Si le protocole Robert était un embryon de coopération européenne, nous regrettons vivement que la France se retrouve isolée, parce qu'elle a retenu une solution peu populaire chez ses voisins.

Concernant la sécurité des données centralisées, je veux bien entendre que d'autres fichiers seraient moins bien protégés, mais je ne sais pas si cela suffit à me rassurer. Je tiens toutefois à saluer la démarche, que vous avez engagée, de soumettre votre solution à Bug Bounty, l'Anssi. Revenons sur la question centrale des libertés fondamentales. Nous sommes peut-être à un tournant de la société : avec la vidéo surveillance, les écoutes téléphoniques et le notre monde est aujourd'hui fondé sur une méfiance généralisée entre les individus. Nous avons aujourd'hui le sentiment d'aller encore plus loin, si ce n'est trop loin : une application dont on ne sait pas si elle sera utile, des drones qui volent sans y être autorisés, des attestations de sortie ... Je connais le contexte sanitaire, mes chers collègues, mais il faut savoir dire stop, et je crains que, avec les collègues de mon groupe, nous ne soyons obligés de dire stop à StopCovid. Certes, l'avis rendu par la CNIL n'a pas été aussi tranché que certains opposants à votre projet l'attendaient. Vous l'utilisez habilement dans vos démonstrations. Pour autant, la CNIL ne vous donne pas de blanc-seing. Elle note que l'application utilisera un service de captcha qui permet de vérifier, lors de l'installation, que l'application est utilisée par un être humain, et que ce service sera dans un premier temps fourni par « un service tiers susceptible « d'entraîner la collecte de données personnelles non prévues dans le décret » ou « des transferts de données hors de l'Union européenne ». La CNIL recommande donc des développements ultérieurs de l'application qui permettent rapidement l'utilisation d'une technologie alternative. En effet, il a été découvert, dans le code source que vous avez continué de rendre public, que c'est bien Google qui fournit l'outil captcha. Je reviendrai sur l'avis de la CNIL. Je souhaiterais maintenant évoquer quelques éléments de comparaison internationale. Je comprends que les choix du Gouvernement

Nous ne pouvons pas savoir si certaines personnes voudront faire fuiter telle ou telle concentration de contacts Bluetooth dans quelques mois. Autre exemple asiatique : à Singapour, pays pourtant discipliné, seuls 20 % des habitants ont téléchargé l'application.

la CNIL précise qu'il faudra évaluer l'efficacité de l'application après son lancement. Mais, monsieur le secrétaire d'État, nous aimerions en être convaincus avant

Surtout, nous ne voulons pas de fausses promesses : votre foi dans la technologie- votre dernier élan rhétorique était éloquent -s'apparente à du « solutionnisme » technologique. Nous sommes admiratifs de la compétence et de la virtuosité technologique de nos scientifiques, de nos centres de recherche, de nos industriels et de nos start-up.

La publication du décret dans un délai raisonnable aurait pu rassurer davantage, en permettant la détection d'éventuelles failles de sécurité. L'expérience de la plateforme APB- Admission post-bac -, avec ses 1 582 violations critiques détectées lors des audits commandés par la Cour des comptes, vient alimenter cette inquiétude.

C'est la raison pour laquelle nous avons accepté de voter l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, nettement plus intrusif que StopCovid. Le Gouvernement s'appuie sur l'avis favorable des épidémiologistes, qui constatent un relâchement de la population. Mais ce constat ne concerne qu'une minorité de personnes, la grande majorité de nos concitoyens ayant compris l'enjeu sanitaire qu'ont révélé les multiples expertises diffusées par les médias, en complément de l'information fournie par l'État. Ce n'est pas en les culpabilisant que nous convaincrons nos concitoyens de consentir au traçage pour éviter une deuxième vague et un reconfinement. La clé de la réussite consiste, à établir la confiance de la population dans la décision publique. C'est pourquoi je me satisfais du suivi qui sera réalisé par le comité de contrôle et de liaison Covid-19, dans un souci de transparence du traitement des données.

Prévoyez-vous un paramétrage pour éviter à un utilisateur de recevoir des notifications récurrentes le conduisant à se faire dépister de manière excessive ? La proportionnalité des atteintes à nos libertés individuelles s'apprécie également en fonction de la sécurité apportée à la préservation de nos données personnelles.

l'architecture centralisée du protocole, vous affirmez que le risque d'une dérive est faible, mais il n'est pas nul. La question a été soulevée dans les États ayant choisi une architecture décentralisée, laissant la France et le Royaume-Uni seuls à privilégier la centralisation. Aucun État, même démocratique, n'est à l'abri d'une dérive et d'un détournement de l'application pour tracer les déplacements des citoyens. StopCovid, reconnaissons-le, apporte des garanties en matière de sécurité anonymisation, volontariat total, caractère temporaire déterminé par décret, exclusion de données sensibles, telles que le recensement des personnes infectées, et des zones dans lesquelles les personnes se sont déplacées, suivi des interactions sociales et non-surveillance du respect des mesures de confinement.

L'infiltration du numérique dans tous les pans de l'administration et de notre vie privée n'est pas sans danger. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire et qu'on a le droit de le faire. Ce n'est pas parce que l'on vous fait visiter une pièce que l'on accepte de vous donner les clés du logement. Pour les innovations numériques comme pour le reste, le facteur humain demeure central en toutes circonstances. La confiance est également un élément incontournable pour garantir l'adéquation des dispositifs à nos principes. Pour conclure, une partie de mon groupe soutiendra la mise en place de StopCovid. Nous nous réjouissons de ce débat qui permet au Parlement, comme c'est son rôle, de se prononcer en toute conscience à un moment aussi important pour nos concitoyens. La parole

soulève une question extrêmement importante : je me réjouis que cette application ait été développée dans un cadre public, parce qu'il ne faut pas laisser

je ne désespère pas de trouver une voie commune avec nos partenaires européens. Comme vous le savez, nous travaillons à un nouveau protocole dénommé Désiré. Une première réunion avec les Italiens, les Espagnols et les Allemands s'est tenue hier au sein de la Commission européenne. Si les choses avancent, nous pourrions peut-être atteindre notre but- je reste encore très prudent -au début du mois de juillet prochain, ce qui serait effectivement une belle victoire pour la construction européenne. Cela nécessitera probablement d'autres discussions avec les Gafam, mais nous n'en sommes pas encore là.

sous la responsabilité de la direction générale de la santé, et, pour ce qui concerne une solution décentralisée, une liste de contacts positifs sur un serveur de Google. Je vous laisse seuls

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

la chronique de cette application, c'est l'histoire du renoncement de votre gouvernement à notre souveraineté numérique. Je prendrai trois exemples. Tout d'abord, je rappelle que la plateforme des données de santé est hébergée par Microsoft.

Isolés en Europe, vous avez échoué à imposer vos choix technologiques à Apple et à Google, et vous subissez ce qu'ils vous imposent. important, pour être efficace, l'application devra être ouverte en permanence pour recevoir des informations du flux Bluetooth. Cette perméabilité continuelle est déconseillée par les constructeurs, il s'agit d'une faille importante de sécurité des terminaux- nous le savons tous ici. L'utilisation de cette application repose sur la confiance : quelles garanties

les garanties apportées en termes de sécurité informatique, comme je l'ai dit, nous prenons toutes les mesures possibles : nous avons par

impossible d'affirmer qu'il n'y a aucune faille : il y en a même dans les plus importants fichiers informatiques, y compris ceux des agences de renseignement. Ce serait un peu présomptueux de ma part de vous dire le contraire s'agissant du fichier StopCovid.

sceaux, madame, monsieur les secrétaires d'État, mes chers collègues, concernant l'application de traçage des cas contacts, la France a fait le choix d'une architecture centralisée. Les informations issues des téléphones remonteront à un serveur, qui sera chargé de les traiter, afin de notifier aux personnes concernées qu'elles ont été en contact avec une personne qui s'est déclarée malade de façon anonyme. Cette solution, également retenue par le Royaume-Uni, a cependant fait l'objet d'une opposition de la part de Google et d'Apple. Ces entreprises, qui détiennent ensemble le monopole des systèmes d'exploitation des smartphones, ont fait pression pour que les applications de traçage utilisent une architecture décentralisée, c'est-à-dire que les informations restent sur les téléphones et ne soient pas stockées sur un serveur centralisé. L'Allemagne, suivie notamment par la Suisse et l'Italie, a accepté de recourir à la solution préconisée par les géants du numérique. Tous les pays européens n'auront donc pas la même structure d'application, au premier rang desquels la France et l'Allemagne. Cette division au sein du couple franco-allemand nous interpelle, car ces applications ont vocation à être utilisées à travers l'Europe, dès que les frontières seront rouvertes, au sein de l'espace Schengen. Monsieur le secrétaire d'État, ma question est double et porte sur ces différences d'architecture : ne seront-elles pas un obstacle à l'interopérabilité des différentes applications nationales ? Par ailleurs, pouvez-vous nous dire quelles sont les différences en matière de cybersécurité ? Y a-t-il une architecture plus vulnérable que l'autre ? La parole

techniques, l'Allemagne a préféré retenir la solution développée par Apple et Google plutôt que la solution française. Je ne vais pas vous mentir : la possibilité que les solutions décentralisées et centralisées soient interopérables est très limitée. Il sera très compliqué d'avoir une solution interopérable au niveau européen, et je le regrette.

c'est que la solution décentralisée est significativement plus facile à attaquer que la solution centralisée. Encore faut-il, dans une démocratie, faire confiance à l'État sur le fait qu'il utilisera bien le serveur central pour ce à quoi il doit servir et pas pour autre chose.

Mes chers collègues, cela fait près d'une heure que nous discutons de l'application StopCovid. Qui est pour ? Qui est contre ? Quel sera son niveau d'efficacité ? Est-elle au point techniquement ?

Dans le dossier StopCovid, vous mettez en avant le fait que nous renonçons à la solution prônée par les Suisses et les Allemands, parce qu'elle a été développée par Google et Apple. Dont acte

Nos deux rapporteurs spéciaux, Loïc Hervé et Dany Wattebled, se sont beaucoup investis sur le dossier. L'impression que j'en retire, c'est que, progressivement, les garanties se sont accumulées

transparence, volontariat, sécurité des données, supervision par une autorité indépendante et, enfin, souveraineté, puisque nous n'avons pas transigé avec la volonté d'un système français ne dépendant pas des Gafam.

contaminées. Le système finit par ressembler étrangement, dans ses potentialités, à ce que l'on a vu à Singapour. Dès lors, je me dis qu'il faut laisser sa chance à ce dispositif,

Corinne Féret, pour le groupe socialiste et républicain. Pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement a décidé de mettre en place un système de traçage des contacts des malades, à l'aide d'une application mobile et, de par sa nature, forcément intrusive dans la vie privée. Je regrette que l'urgence que nous ressentons tous, collectivement, face à la crise sanitaire actuelle fasse oublier que le numérique doit être au service de chaque citoyen, qu'il ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Dans ce contexte, il est légitime de s'interroger sur l'opportunité de lancer l'application StopCovid, alors même que nous connaissons un début de baisse et que nous ne pratiquons toujours pas une politique massive de tests. Et c'est sans compter que les Français les plus affectés, les plus fragiles, en l'espèce les plus âgés, sont aussi les moins sensibilisés aux nouvelles technologies et aux applications téléchargeables sur téléphone portable. De plus, alors que 77 % des Français possèdent un smartphone, il faudrait que plus de 80 % de la population utilisent l'application pour qu'elle soit efficace. Vous reconnaissez vous-même, monsieur le secrétaire d'État, qu'il y a une incertitude technologique Dans ces conditions, il serait préférable d'admettre que l'application StopCovid présente un intérêt limité dans la lutte contre le Covid-19 et, surtout, qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée aux droits et libertés des citoyens. Je souhaite aussi insister sur la situation particulière des mineurs équipés de smartphone, qui pourront, demain, télécharger l'application. Comme le rappelle la CNIL dans son avis rendu hier, il conviendra de veiller au contenu de l'information diffusée et de s'assurer que StopCovid soit utilisée à bon escient que le message d'alerte susceptible d'être adressé à ces adolescents soit adapté et bien interprété. Ma question est donc la suivante : monsieur le secrétaire d'État, avez-vous prévu que soient intégrés, dans l'information fournie aux utilisateurs, des développements spécifiques, à la fois pour les mineurs adolescents et pour leurs parents ?

Au détour de la dramatique crise sanitaire du Covid-19, le numérique entre à grands pas dans le monde de la santé. En particulier, le projet d'une application de traçage des personnes touchées par le virus a suscité de nombreuses réflexions et discussions publiques. Le Gouvernement a finalement décidé de lancer l'outil StopCovid, dont nous parlons ce soir, pour compléter sa politique de lutte contre la propagation de l'épidémie. Je ne reviendrai pas sur la question de la protection des données, si ce n'est pour rappeler que mon groupe, souligné Françoise Laborde, est bien entendu attaché au respect des libertés individuelles et qu'il prend acte des dernières recommandations de la CNIL, en particulier sur les précautions à renforcer

Apple ne permettant pas l'accès au Bluetooth en continu en arrière-plan d'une application, l'outil StopCovid ne pourrait pas, semble-t-il, être utilisé sur un iPhone.

Par ailleurs, quel impact aura l'application, si elle reste ouverte à l'arrière-plan, sur la batterie du téléphone ? La parole est à M.

avec l'appui de nombreux industriels qui s'investissent dans notre pays. Vous avez fait le choix de recourir à notre savoir-faire national pour le mettre au service de l'intérêt général et du progrès humain, dans un domaine où l'on excelle souvent trop discrètement. Vous avez parlé de panache ... Ma moustache en a frémi À ce jour, les tests ont été menés sur les 100 références de téléphone les plus utilisées par les Français, de 17 marques différentes. Les tests ont démontré que l'application fonctionnait de manière très satisfaisante sur l'ensemble des modèles du parc de référence. Pour autant, près de 23 % des Français ne disposent pas de smartphone ou ne sont pas à l'aise avec le numérique. Or, le virus n'a pas de frontière et touche toutes les classes sociales. Ce public, dont il n'est pas imaginable qu'il puisse être exclu du processus, désire souvent être acteur dans le combat contre le Covid-19. C'est pourquoi de nombreuses entreprises françaises se sont investies dans la recherche et le développement de produits innovants, pouvant répondre à cette attente. Je pourrai par exemple citer Sigfox, une société toulousaine spécialiste des réseaux de télécommunication bas débit, qui travaille à un prototype de bracelet connecté indépendant de Google et d'Apple. La France, comme d'autres pays, d'ailleurs, ne ferme pas la porte à la solution du bracelet connecté pour des tiers dépourvus de smartphone, à l'instar des personnes âgées, bien sûr, ou des personnes modestes. Le Gouvernement doit pouvoir proposer des solutions à ces publics, pour qu'ils soient eux aussi en mesure, sur la base du volontariat, de compléter l'action des médecins et de l'assurance maladie. Monsieur le secrétaire d'État, à ce jour, l'option d'un bracelet connecté est-elle toujours envisagée ? D'autres choix de ce type sont-ils à l'étude pour favoriser la participation bénévole de ces Français, éloignés des objets connectés ? Si oui, l'État entend-il contribuer à la distribution de ces outils ? La parole est à M. le secrétaire

Je tiens tout d'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet : les rapporteurs, mais aussi les orateurs, qui nous ont parfaitement expliqué les enjeux du débat. Après avoir écouté les uns les autres, ce n'est pas tant le danger de l'application StopCovid qui m'inquiète le plus ; c'est son efficacité Il faut considérer cette application à sa juste mesure. Il serait paradoxal, à mon sens, d'être plus exigeant en termes de données personnelles avec StopCovid qu'avec les Gafam.

que sur la lutte contre le Covid-19. Toutefois, mes chers collègues, même si certains indicateurs peuvent sembler rassurants, la maladie rôde toujours ! Elle menace encore les plus fragiles, ceux d'entre nous qui risquent leur vie. Rappelons que nous ne disposons, pour l'heure, ni d'un vaccin ni d'un traitement, et nous n'avons pas non plus l'assurance d'en disposer très prochainement. Faudrait-il rester passifs et ne compter que sur le confinement, avec son cortège de drames économiques et sociaux, pour lutter contre la maladie ou son éventuel retour ? Je m'étais exprimé en ce sens lors du débat sur les brigades anti-Covid. Je persiste et signe : nous n'avons pas d'autres moyens de lutter contre la maladie que de tester, tracer et isoler. Si l'application StopCovid y participe, tant mieux

est possédée par plus de 60 % de la population française. Une seule ! Mon objectif n'est certainement pas d'atteindre ce niveau. Par ailleurs, une couverture de 60 % de la population française n'aurait pas beaucoup de sens, puisque nous réfléchissons en termes de bassin de vie. Donc, si une ville est couverte,

Pendant plusieurs semaines, les Français ont été enfermés chez eux, privés de leur liberté fondamentale d'aller et de venir. Pendant plusieurs semaines, notre pays a lutté, à l'aveugle, contre l'épidémie de Covid-19. Voilà un mois, le triptyque « protéger, tester, isoler » a guidé les conditions de notre liberté, pour partie retrouvée. Il consiste à passer de la lutte à l'aveugle à la lutte informée. Notre stratégie a été largement guidée par les capacités disponibles en équipements de protection, en tests, en applications. Aucune de ces capacités ne suffit à elle seule, mais toutes sont nécessaires, je le vu la connaissance que nous avons actuellement du virus, peut-être encore insuffisantes. D'autres pays ont procédé autrement. Je pense à la Corée du Sud, qui, instruite par des épidémies précédentes, a misé sur la connaissance la plus fine possible de la propagation du virus et sur l'information de la population. Si nous n'avons pas été prêts, monsieur le secrétaire d'État, pour cette épidémie, il n'est pas interdit de l'être pour la prochaine L'application StopCovid testée en grandeur nature pourrait servir à nouveau face à une maladie encore plus insidieuse et à la létalité encore plus élevée. Si nous n'avons pas été prêts pour cette épidémie, d'autres le seront, avec moins de garanties pour nos données de santé, nos libertés et notre souveraineté, comme l'ont souligné Philippe Bas et Bruno Retailleau. Pour informer plutôt que d'enfermer, je suis favorable à l'usage d'une application raisonnée, maîtrisée, avec des garanties publiques et individuelles. Je m'interroge toutefois sur un point-

recourir à une application de suivi des contacts rapprochés est un choix très discutable. Sur le plan de l'efficacité, tout d'abord, la théorie pure et parfaite sur laquelle se fonde application est, indépendamment même de la question du volontariat, difficilement transposable à la réalité des Français

la génération de données de santé en transit dans le comporte un risque important de vol de ces données. Ce sont la vie privée des utilisateurs et leurs données personnelles et de santé qui sont en jeu ! Le piratage n'est pas une vue de l'esprit : à n'en pas douter, toutes ces données suscitent d'ores et déjà

pour diverses personnes, voire des États. Au passage, nous aurons aussi abandonné une part de liberté. Vous savez ce que disait Benjamin Franklin à ce sujet : « Un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. En prime, nous aurons gagné une ambiance de défiance généralisée ... Ne faudrait-il pas plutôt parier sur la confiance, une confiance réciproque qui s'est un peu perdue ces derniers temps ? temps ? Comme l'explique l'historien Noah Harari, « une population informée et motivée est beaucoup plus puissante et efficace qu'une population ignorante et contrôlée par la police ».

du débat, mais essentiel, car il souligne la potentielle impuissance de l'État dans le monde numérique. Dans la genèse de l'application StopCovid, le Gouvernement s'est heurté au refus des deux géants Apple et Google de lever certaines barrières techniques sur leur système d'exploitation. Vous avez trouvé une astuce, mais admettez, monsieur le secrétaire d'État, que c'est inadmissible ! En réalité, la puissance publique s'est retrouvée dans la position de n'importe quel développeur d'applications face au duopole Apple-Google, qui impose ses conditions sans se justifier et de façon opaque. Cette situation est d'autant moins acceptable qu'elle aurait pu être prévenue, si un principe de neutralité des smartphones avait été consacré, comme le Sénat l'avait proposé en adoptant une proposition de loi de la commission des affaires économiques, votée à l'unanimité des groupes politiques de notre assemblée le 19 février dernier. Monsieur le secrétaire d'État, cette crise sans précédent doit être l'occasion de tirer des enseignements et des leçons pour l'avenir et de mettre fin aux errements du passé.

Sur le fond, vous avez raison : ce qui s'est passé est inadmissible. De fait, aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens juridiques de contraindre Apple et Google à modifier leur attitude dans ce qui s'apparenterait, si nous étions dans le champ commercial, à un abus de position dominante. C'est à peu près de

que cette expérience apporte de l'eau au moulin de tous ceux, dont vous faites partie, qui dénoncent une situation oligopolistique et un marché fermé sur des infrastructures qui pourraient s'apparenter à des infrastructures essentielles.

à l'article 56 du règlement ; aucune explication de vote n'est admise.